Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, attentat après attentat, nous avons l'impression de répéter les mêmes mots, d'assister aux mêmes cérémonies, de rencontrer les mêmes familles dévastées par le chagrin. Pourtant, ce qui s'est passé à Rambouillet, le 23 avril dernier, a constitué pour la communauté de la police et pour les Rambolitains un degré supplémentaire dans la douleur que nous avons déjà vécue. Cet attentat a touché dans ce commissariat des femmes et des hommes qui, pour beaucoup d'entre nous, et pour moi-même, sont familiers. Cet islamiste a assassiné Stéphanie Monfermé, que nous connaissions particulièrement. Ce crime a été pour tous les Yvelinois, après Magnanville et Conflans-Sainte-Honorine, la nouvelle étape d'une tragédie qui paraît ne jamais finir. Aucun lieu de notre territoire n'est désormais épargné par l'islamisme radical. Notre seule volonté doit être l'efficacité dans la lutte contre ce terrorisme et dans la protection de nos concitoyens. Face à ce que certains qualifient de « guerre », face à la volonté de diviser notre nation par cette violence, ne cédons pas. Répondons avec détermination, en démocrates solides sur nos valeurs. C'est ce que nous avons réaffirmé à vos côtés, monsieur le Premier ministre, et aux côtés des élus présents vendredi dernier. Soyons déterminés, c'est notre responsabilité

jeudi dernier, le Président de la République a annoncé la mise en place d'un pass sanitaire pour concilier sortie de crise et respect des libertés individuelles. La vaccination n'étant pas encore accessible à tous et restant facultative, l'idée de mettre en place un passeport vaccinal a été écartée au profit d'un dispositif moins restrictif. Le pass sanitaire sera donc délivré sur présentation d'une attestation vaccinale, d'un certificat de guérison ou du résultat négatif d'un test PCR ou antigénique réalisé dans les Il devrait être obligatoire dès le 9 juin dans les lieux particulièrement fréquentés, tels que les foires et les salons, et à partir du 30 juin pour participer à des rassemblements de plus de 1 000 personnes. Ce pass sera également un prérequis pour l'accueil des touristes étrangers. Dans l'attente du prochain débat au Parlement à ce sujet, plusieurs questions restent en suspens. Pour l'heure, l'Agence européenne du médicament a reconnu quatre vaccins : Pfizer, AstraZeneca, Moderna et Johnson & Johnson. la suivante : d'autres vaccins seront-ils acceptés par le dispositif pour permettre, par exemple, d'accueillir des touristes de pays ayant fait un choix vaccinal différent du nôtre ? Nous aimerions également savoir si le pass sanitaire sera obligatoire pour les mineurs et, le cas échéant, à partir de quel âge. À l'échelon européen, un cadre commun est en cours de définition les eurodéputés se sont prononcés, le 29 avril dernier, sur la mise en place d'un certificat vert numérique d'ici à la fin du mois de juin. Son instauration devrait permettre de faciliter les déplacements entre les pays membres. Pourriez-vous nous confirmer que sa délivrance se fera dans les mêmes conditions que le pass sanitaire ? Enfin, pouvez-vous nous éclairer sur les conditions de la levée des mesures de quarantaine ?

Tout d'abord, je salue la résilience des Français dans cette crise sanitaire, ainsi que leur engouement pour la vaccination. Près de 16 millions de Français ont reçu au moins une dose, soit 30 % de la population.

PCR, les tests positifs de moins de trois mois, ainsi que les certificats de vaccination. La vaccination étant fortement encouragée, le pass sanitaire ne pénalisera pas les personnes non vaccinées contre la covid-19, d'autant que, je le rappelle, les tests sont gratuits en France, ce qui est la mise en place d'un certificat sanitaire permettant aux citoyens européens de voyager au sein de l'Union européenne est en train d'être débattue. Plusieurs compagnies aériennes envisagent également d'utiliser ces passeports sanitaires pour les vols hors de France. Ces éléments sont actuellement discutés

Madame la ministre, voilà maintenant plus de deux mois que l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, l'AP-HM, est dans l'attente d'un nouveau directeur général. de deux mois que l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille, l'AP-HM, est dans l'attente d'un nouveau directeur général. Les procédures ont pourtant été respectées de façon scrupuleuse. Un consensus local a même été établi concernant les candidatures proposées par la présidente du conseil de surveillance, Mme Rubirola, le doyen de la faculté de médecine, le professeur Leonetti, par ailleurs conseiller régional, et le président de la commission médicale d'établissement, la CME, le professeur Rossi. Cette situation est d'autant plus pénalisante que, dans le cadre du Ségur de la santé, les autres CHU ont pris l'initiative de proposer des plans de financement complémentaires, récemment acceptés par les tutelles. Malheureusement, à Marseille, du fait de la situation bloquée, aucune initiative n'a été prise en ce sens, privant ainsi cette institution d'un financement complémentaire absolument nécessaire. l'incompréhension est totale face à cette situation, et le ressenti est celui d'un certain mépris pour les acteurs de terrain. Ce sentiment de mépris est exacerbé- c'est un doux euphémisme -par la rumeur entretenue par la presse selon laquelle le nouveau directeur de l'AP-HM pourrait être M. Salomon, actuel directeur général de la santé, décision prise par Paris, sans tenir compte du choix des décideurs locaux, dont Renaud Muselier, qui étaient tous d'accord sur la personne de M. Crémieux. Madame la ministre, pouvez-vous nous indiquer quelle est votre décision quant à la nomination du nouveau directeur de l'AP-HM ? La

à la tête de cet ensemble si prestigieux. Je puis vous confirmer que le processus de recrutement a été lancé, comme vous l'avez souligné. Les candidatures ont été examinées par un comité de sélection locale, avec, d'une part, l'agence régionale de le président de la commission médicale d'établissement et la mairie de Marseille. Trois noms ont été proposés au ministère. À l'issue de ce processus, les échanges se sont poursuivis, notamment avec les acteurs locaux. Deux éléments importants justifient la poursuite des discussions. Compte tenu de l'importance de ce centre et de la difficulté de diriger une telle institution, le processus de désignation est capital : il est normal d'en prendre le plus grand soin,

Madame la ministre, la direction générale des collectivités locales vient de publier la répartition de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, pour l'année 2021.

Ces baisses ne concernent qu'un tiers des communes de plus de 20 000 habitants, mais elles touchent 55 % des communes de moins de 1 000 habitants. Ces communes, qui ont déjà une dotation forfaitaire par habitant bien inférieure à celle des communes urbaines, observent ainsi leurs recettes, déjà limitées, diminuer d'année en année, et éprouvent de plus en plus de difficultés à équilibrer leur budget. Que les communes de toutes tailles ignorent les causes de ces diminutions, tant le calcul de la DGF est opaque, accentue l'incompréhension des élus concernés.

traduit le fait que les charges d'une commune croissent avec sa population. Cette corrélation n'est contestée par personne, pas même par ceux qui avaient envisagé une réforme de la DGF. Pour prendre un exemple que vous connaissez bien, monsieur le sénateur, la commune de Bernay reçoit 250 euros de DGF par habitant, contre 172 euros en moyenne pour les communes de son intercommunalité. Pourquoi ? Tout simplement parce que Bernay est au coeur d'un bassin de vie et fournit des services et des équipements à une population qui dépasse largement son territoire. J'ajoute qu'il faut envisager la question dans une perspective dynamique. Depuis 2017, les communes de moins de 3 500 habitants ont gagné 72 millions d'euros de DGF, quand, sous le quinquennat précédent, elles avaient perdu 700 millions d'euros de dotation.

À l'heure où de très nombreuses familles sont confrontées à la précarité, des associations demandent le prolongement de la trêve hivernale jusqu'au 31 octobre. En effet, les expulsions locatives, déjà en hausse constante depuis des années, pourraient doubler cette année si rien n'est fait. Selon l'Insee, parmi les 10 % de ménages les plus modestes, 35 % ont subi une dégradation de leur situation financière. La Banque de France prévoit, elle, un pic du chômage supérieur à 11,5 % d'ici à quelques mois. Comme le souligne la Confédération nationale du logement, qui a lancé une pétition à ce sujet, il convient de ne pas ajouter à la situation économique et psychologique dramatique l'angoisse d'une expulsion pour des milliers de ménages. Une expulsion locative n'est pas un simple acte administratif ; c'est un drame humain aux multiples répercussions. C'est la raison pour laquelle nous soutenons soutenons l'idée d'une « sécurité sociale du logement », un fonds de solidarité nationale. Madame la ministre, que comptez-vous faire pour garantir le droit au logement, reconnu comme un objectif à valeur constitutionnelle ? Allez-vous, enfin, reporter la trêve hivernale,

face à la crise sanitaire que nous connaissons, nous avons pris des mesures exceptionnelles pour protéger les locataires vulnérables. Dès l'année dernière, à l'issue de la trêve hivernale, que nous avons prolongée jusqu'à juillet 2020, nous avons fixé comme consigne qu'il n'y ait pas d'expulsion sans proposition de relogement ou d'hébergement, consigne qui s'est traduite par un nombre d'expulsions exceptionnellement bas en 2020. Nous prolongeons de nouveau la trêve hivernale cette année, du 31 mars au 31 mai. Nous avons par ailleurs ouvert un nombre exceptionnel de places d'hébergement pour la mise à l'abri. Nous en sommes aujourd'hui à plus de 200 000 places. C'est un geste de solidarité très fort vis-à-vis des personnes en difficulté. Nous devons désormais réussir la fin de la trêve, la fin de ces mesures temporaires, pour assurer un retour progressif au cadre de la loi. Nous préparons donc depuis plusieurs mois, avec toutes les associations de solidarité, la fin de cette trêve, avec une priorité : continuer à protéger les personnes précaires et vulnérables. Si une expulsion a lieu après le 1 juin, elle sera assortie d'une proposition de relogement ou,, d'hébergement. Un travail sera réalisé également en amont de l'expulsion, pour proposer un accompagnement social et une solution aux locataires. cette transition face au droit commun, car nous devons aussi prendre en compte la situation des petits propriétaires, dont le loyer constitue une source importante de revenu. Nous ne pouvons pas avoir une année blanche en matière d'expulsions. C'est aussi pour cette raison que l'État s'est engagé à indemniser rapidement les propriétaires concernés. Nous abonderons dès juillet prochain le fonds d'indemnisation des propriétaires bailleurs d'un montant complémentaire, estimé à 20 millions d'euros. Enfin, nous avons décidé de mettre en place à titre exceptionnel pour 2021 quelque 30 millions d'euros de fonds d'aide aux impayés de loyers. Il s'agit d'une demande portée par les associations. Cette somme viendra abonder les fonds solidarité logement des collectivités locales pour aider les ménages en difficulté à se maintenir dans leur logement. Madame la ministre, votre réponse est loin de me satisfaire. Il faut sortir le logement de la logique marchande. Nous avons besoin de moyens financiers non seulement pour le fonds d'indemnisation, mais aussi pour les bailleurs, afin de construire du logement social et pour la réquisition des logements vacants. Ce ne sont pas vos vagues instructions aux préfets ni vos annonces qui changeront la donne. Et permettez-moi de vous rappeler que des solutions d'hébergement ne seront jamais équivalentes à un accès pérenne au logement. logement. La parole est à Mme Nadège Havet, pour le groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'éducation nationale. Mes premiers mots vont aux équipes pédagogiques et aux élèves qui, partout en France, ont repris le chemin de l'école lundi dernier.

Nos terminales, notamment, abordent la dernière ligne droite avant ce rite de passage que constitue toujours le baccalauréat, un diplôme cadre qui est aussi une entrée dans l'enseignement supérieur et dans l'âge adulte. Des diplômes, des épreuves, Des diplômes, des épreuves, le stress qui va avec ... Un stress accru dans la période actuelle. Les épreuves, le grand oral et la philosophie arrivent. Certains expriment des doutes quant à la faisabilité pour les lycéennes et lycéens de plancher en présentiel. Des inégalités dans l'avancement dans les programmes, en fonction des établissements, sont mises en avant. Nous le savons, le virus a frappé partout, mais il n'a pas touché tous les territoires et tous les lycées de la même façon, ni avec la même intensité et les mêmes conséquences en matière de continuité pédagogique. Même si la France a connu un maintien du nombre de jours d'école remarquable par rapport aux autres pays depuis le début de la pandémie, face à ces constats, monsieur le ministre, faut-il prévoir un contrôle continu généralisé ? Faut-il envisager des aménagements supplémentaires ? Certains ont déjà été opérés : je pense aux épreuves de spécialité de mars dernier, aux épreuves anticipées de français de la classe de première et au contenu de l'épreuve de philosophie. et au contenu de l'épreuve de philosophie. Vous avez rencontré hier les syndicats et les organisations lycéennes, afin d'étudier de nouvelles pistes pour ajuster les épreuves. Pourriez-vous nous en dire plus ? En particulier, des élèves inscrits dans les écoles hors contrats ? La parole

du baccalauréat. Nous disposons également d'un comité de suivi spécifique de la voie professionnelle. Qu'il s'agisse du baccalauréat général et technologique ou du baccalauréat professionnel, nous nous adaptons. Vous avez relevé les plus importantes de ces adaptations récentes, notamment le fait d'avoir transformé en contrôle continu des épreuves terminales qui étaient prévues en mars dernier. Nous avons encore devant nous pour le baccalauréat général et technologique l'épreuve de philosophie écrite et le grand oral. Comme vous l'avez souligné, j'ai échangé hier, par visioconférence, avec les organisations lycéennes. Nous discutons aussi avec les organisations représentatives des personnels.

jours. La parole est à M. Franck Montaugé, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Monsieur le président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre, que je salue. Des politiques dures pour les faibles et faibles pour les forts votre réforme de l'assurance chômage, comme un marqueur politique de plus, montre que vous n'avez pas le souci des situations de vie problématiques que subissent au quotidien beaucoup trop de nos concitoyens. Le chômage, ce n'est pas un concept théorique, c'est une réalité humaine dévastatrice que je connais personnellement, dans la chair de ma chair ! C'est un cancer sociétal, qui plonge des femmes et des hommes responsables, désireux de travailler, attachés, quoi qu'en disent honteusement certains, à leur contribution économique à la société française, en même temps qu'à leur autonomie de vie. Je crois que vous ne savez pas ce que c'est moralement que de se retrouver proche de la fin de ses droits, quand on a de jeunes enfants et souvent une maison qu'il va falloir vendre, parce que le projet de vie vole en éclats à cause de la perte d'emploi Moi, comme des millions de Français, je le sais. Et votre politique n'en apparaît que plus injuste et violente, dans cette période où les problèmes sociaux et sociétaux sont, hélas, déjà là, et devraient encore Faire payer aux plus faibles d'entre nous près de 1,5 milliard d'euros à un moment où, à bon droit, on inonde l'économie de centaines de milliards d'euros, il fallait oser, et vous l'avez fait Ma question est simple : comment envisagez-vous de traiter ce dossier à l'avantage des chômeurs, qui ne demandent qu'à retrouver au plus vite un travail utile, sensé, à la hauteur de leur qualification et au bénéfice de notre société ?

est injuste. Un demandeur d'emploi travaillant à mi-temps perçoit une allocation très inférieure à celle que toucherait un demandeur ayant travaillé une semaine sur deux pour le même salaire et le même nombre d'heures travaillées. Cela n'est pas satisfaisant. Par ailleurs, le système est coûteux. L'alternance entre contrats courts et et périodes de chômage coûte environ 3 milliards d'euros par an à l'assurance chômage. Plus globalement, le régime est déficitaire depuis plus de dix ans, avec près de 40 milliards d'euros de dettes cumulées avant même la crise de la covid. Le système actuel a enfermé de nombreux demandeurs d'emploi dans le chômage, et il a encouragé la précarité. J'en veux pour preuve un seul chiffre le nombre de CDD de moins d'un mois a augmenté de 250 % en dix ans. Vous avez tout fait pour ! Avec le bonus-malus, les entreprises seront désormais incitées à proposer davantage de CDI et à allonger la durée des CDD.

et son déploiement sera progressif. Je veux rassurer nos concitoyens : notre système d'assurance chômage restera très protecteur, puisque nous maintenons une durée longue d'indemnisation, un taux de remplacement relativement élevé et des conditions d'affiliation très ouvertes. Enfin, le montant global d'indemnisation du demandeur d'emploi restera le même ; c'est la durée d'indemnisation qui est prolongée par la réforme. La parole la ministre. Monsieur le Premier ministre, le « quoi qu'il en coûte » s'est iniquement et cyniquement transformé en un « quoi qu'il en coûte socialement ». Quant à nous, nous le rejetons. Nous combattrons avec fermeté et avec sens de la justice cette politique de décohésion sociale,

durant la période estivale, nos communes vivent au rythme des fêtes locales et des bals populaires, tout particulièrement dans le sud de la France. Cette tradition a été interrompue l'été dernier en raison de la crise sanitaire, et, cette année, tous les acteurs s'interrogent sur la possibilité de retrouver ces moments forts de convivialité. Les musiciens souhaitent retrouver leur pupitre après une année noire. Les organisateurs, qu'il s'agisse des communes ou des associations, ne connaissent pas encore, à ce jour, les protocoles sanitaires et les jauges qu'ils vont devoir respecter. Les fêtes estivales de plein air sont traditionnellement gratuites et, le plus souvent, organisées par des comités des fêtes ou des associations de proximité : ceux-ci mettent en place des buvettes, qui sont une source de revenus non négligeable lors de ces rassemblements de population. Aussi, à quelques semaines de l'été et dans la perspective du prochain déconfinement annoncé, les musiciens n'attendent qu'une chose : pouvoir jouer et se produire à nouveau dans ces fêtes locales. Car il n'y a pas que les grands festivals pour animer nos territoires. Je n'oublierai pas non plus la situation des forains, qui attendent avec impatience de pouvoir installer leurs manèges ou autres attractions. Madame la ministre, en 2020, les normes sanitaires entraînaient l'impossibilité d'organiser de tels événements. Pouvez-vous nous indiquer si, pour l'été qui arrive, les fêtes locales et autres manifestations populaires de plein air pourront reprendre, sans que des protocoles sanitaires excessifs fassent peser une responsabilité insoutenable sur les épaules des organisateurs

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Christian Bilhac, vous avez souligné l'importance, aux côtés des manifestations culturelles classiques,

Je veux être très claire et précise : même si nous avons un calendrier d'élargissement des jauges, des plafonds et de l'heure du couvre-feu, avec des mesures qui seront pratiquement toutes levées

y compris dans les fêtes de village. Ce sont non pas des mesures barrières, parce qu'elles ne nous éloignent pas les uns des autres, mais des mesures de protection. Porter un masque, se laver les mains, respecter les distanciations sociales, c'est du respect ! C'est comme cela que nous arriverons à retrouver une vie normale. Très bien ! La parole La parole est à M. Thomas Dossus, pour le groupe Écologiste - Solidarité et territoires. aux islamo-gauchistes », reprenant le vocabulaire en vogue au Gouvernement. Le 17 avril, un ancien ami du Président de la République, Philippe de Villiers, appelait dans à l'insurrection, pour « éviter la disparition de la France ». Le 21 avril, des généraux ont publié une tribune factieuse, menaçant le pays de guerre civile pour lutter contre « l'indigénisme » et « les hordes de banlieue et n'entraînant que des réactions tardives et timorées de votre gouvernement. Ces actes et propos ne sont pas isolés. Partout, la parole se libère et l'extrême droite la plus radicale passe aux actes. Cette extrême droite est une menace grandissante et mortelle pour notre République. Face à ce danger, les digues ont sauté, avec La République En Marche, qui trouve parfois l'extrême droite trop molle, mais aussi avec une partie de la droite républicaine présente dans cet hémicycle. J'en veux pour preuve la liste interminable d'amendements stigmatisants qui ont été adoptés par le Sénat lors de l'examen du projet de loi « Séparatisme », à l'encontre de nos concitoyens musulmans, ou encore les attaques frontales et scandaleuses de certains ministres ou parlementaires de votre majorité à l'encontre du monde universitaire, qualifié d'islamo-gauchiste. Ces discours ne sont pas sans conséquence, jusque dans nos territoires, notamment à Lyon. dernier, le Gouvernement a annoncé la dissolution du mouvement fasciste Génération identitaire. Cette décision était nécessaire et bienvenue. Ce mouvement est très implanté à Lyon. Dans cette ville, depuis cette dissolution, : le 19 mars, une quarantaine d'hommes ont lancé des pavés et saccagé la vitrine d'une librairie ; le 24 avril, une quarantaine d'individus d'extrême droite ont lancé des projectiles sur une manifestation ; enfin, le 1 mai, le local d'une radio lyonnaise a été attaqué par une quarantaine

votre gouvernement va-t-il cesser d'être complaisant avec l'extrême droite et va-t-il lutter réellement contre son expansion, avec une détermination à la hauteur de la menace qu'elle fait peser sur la République ? Mes

quel qu'il soit, malgré ce que certains élus ont l'air de penser ; un militaire n'est pas un militant ; les armées sont là pour protéger les Français, tous les Français. Quiconque aurait un avis différent déshonorerait nos armées et notre République. Florence Parly a eu l'occasion de l'indiquer, les 52 officiers généraux qui ne sont plus en activité seront traduits devant un conseil supérieur d'armée en vue de leur radiation et les 18 militaires d'active ayant violé le devoir de réserve seront soumis à des sanctions disciplinaires,

le ministre a engagé la procédure de dissolution de Génération identitaire. Le Conseil d'État a estimé que cette association était bien responsable de provocation à la haine et à la discrimination.

Cette hausse de la fiscalité est la conséquence des baisses de dotations et de recettes que les collectivités locales subissent depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et qui ne sont jamais intégralement compensées. C'est aussi la résultante de l'accumulation des dépenses exceptionnelles auxquelles les collectivités locales font face depuis dix-huit mois pour répondre aux besoins de leurs populations, des acteurs économiques et du monde associatif.

Madame la sénatrice Sabine Drexler, vous m'interrogez sur la prise en charge de l'effort budgétaire des collectivités pour la mise en

les ARS, peut et doit être mobilisé pour participer aux dépenses de fonctionnement des centres de vaccination, dans une logique de partenariat entre l'État et les collectivités. Des conventions de subvention sont à cet effet signées entre les ARS et les structures portant les centres de vaccination : elles visent à financer les surcoûts auxquels les collectivités qui mettent en place ces centres sont exposées. Vous le voyez, la réponse est claire. Nous avons affecté, dès le 18 février 60 millions d'euros aux ARS pour les FIR, afin de financer les dépenses les plus urgentes des 1 200 centres ouverts sur le territoire. Ces subventions peuvent comprendre la prise en charge de moyens de fonctionnement, tels que le secrétariat, la coordination, l'accueil, ainsi que la mobilisation des agents pour le fonctionnement des centres le week-end, en plus de leur temps de travail habituel, ce qui peut être aussi considéré comme un surcoût et donner lieu à un financement. Le recrutement de personnes complémentaires peut également donner lieu à un financement. aux personnels prescripteurs, effecteurs, indemnisés par la sécurité sociale ou à la participation des sapeurs-pompiers, qui peut également être prise en charge dans certaines conditions.

Madame la ministre, les communes se sont fortement investies en cette période inédite, et elles ont une nouvelle fois montré leur réactivité et leur implication. les dotations forfaitaires promises par le Gouvernement sont largement insuffisantes. La situation financière des collectivités locales se dégrade plus vite que vous ne le pensez. Les budgets dits « covid » pèsent extrêmement lourd. Les collectivités ne pourront pas continuer à faire toujours plus de dépenses avec toujours moins de rentrées d'argent. Votre gouvernement a fait des promesses pour que la prise en charge soit bien supérieure. Les élus locaux attendent que vous les respectiez.

Monsieur le Premier ministre, le monde traverse la plus grande crise sanitaire de la période moderne. Si nous disposons aujourd'hui de vaccins contre le covid-19, nous faisons face à une vague plus violente encore que les précédentes. Nous devons accélérer le rythme de vaccination partout, à l'échelle de la planète, y compris en France. Nous ne sommes toutefois pas convaincus que la stratégie européenne et mondiale se donne tous les moyens d'y parvenir. Plus de cent gouvernements nationaux, dont l'Inde et l'Afrique du Sud, avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et de nombreux experts de santé, plaident pour une dérogation temporaire aux règles de propriété intellectuelle, afin de permettre une couverture vaccinale la plus large possible.

Selon, la plupart des habitants des pays africains ne seront pas vaccinés avant 2023, et il faudra attendre 2022 pour ceux de nombreux pays émergents. Combien de nouveaux variants d'ici là ? Combien de morts supplémentaires ? Combien d'économies à terre ? Monsieur le Premier ministre, les vaccins contre le covid-19 doivent devenir un bien commun de l'humanité. Ma question est donc simple : la France va-t-elle porter la levée temporaire des règles de propriété intellectuelle pour ces vaccins en Europe et dans le monde ?

la France a pris la tête d'un certain nombre de pays développés, qui sont de grands acheteurs de vaccins, pour fournir, notamment aux pays du Sud, des doses de vaccin. Je pense aux centaines de milliers de doses qui ont été données unilatéralement par la France dans le cadre de l'initiative

parce que ce n'est pas un problème de brevet. Même si tous les brevets étaient en accès libre, il n'y aurait pas de production supplémentaire pour les pays du Sud avant la fin de 2022, compte tenu de la complexité industrielle que cela représente. Il faut en effet pour « valider » une usine. Ensuite, il est nécessaire que les industriels continuent à investir dans la recherche pour développer des réponses aux nouveaux variants. Si nous leur retirons la propriété intellectuelle, ils risquent

Chaque mois, le groupe américain Bloomberg établit un classement de la résilience des 53 économies les plus importantes. Singapour est en tête de ce classement. Très loin derrière, la France se situe en 42 position ; 16 États européens sont mieux classés que nous. pays a perdu 18 places par rapport au mois précédent. Cela s'expliquerait par l'arrivée des variants et l'échec des « mesures de freinage ». La campagne vaccinale de 2009 pour la grippe H1N1 avait eu le mérite de ne laisser aucun de nos compatriotes résidant à l'étranger sur le bord du chemin. Ce n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. On ne saurait remettre en cause le sérieux des dix critères de ce classement, qui prend en compte non seulement des indicateurs de la propagation de la covid, mais aussi la qualité de vie. Ces critères sont notamment le nombre de cas et le taux de mortalité au cours du dernier mois, le nombre de décès depuis le début de la pandémie et la part de la population couverte par les vaccins. Pour ce qui est de la qualité de vie, sont notés la sévérité du confinement, la variation du produit intérieur brut, la couverture universelle des soins de santé et l'indice de développement humain. À titre d'exemple, avec 1 609 morts pour 100 000 personnes, la France est le troisième plus mauvais élève dans le classement Bloomberg. Nul ne mettra en doute des sources qui sont, pour n'en citer que trois, l'université d'Oxford, le Fonds monétaire international et Google. Monsieur le Premier ministre, le Gouvernement semble satisfait de son action, alors que les résultats ne sont manifestement pas au rendez-vous. Comment expliquez-vous une telle contre-performance ?

Ce même classement dit aussi que la France est un pays où les habitants ont un bon accès à la vaccination. Les résultats sont là, et ce sont des faits, madame la sénatrice.

collectivement saluer, de nos soignants, et parce que nos concitoyens respectent les mesures sanitaires que nous avons dû prendre. La situation est en train de s'améliorer, et je pense qu'il serait de bon ton de le saluer. La parole est à Mme Madame la ministre, je ne suis pas surprise de votre réponse. Vous avez pourtant une belle marge de progression. Ce classement n'est pas un cas isolé, puisque l'indice de performance covid développé par l'Institut Lowy de Sydney nous classe 71 sur 102 pays au mois de mars, ce qui n'est guère mieux Pour l'instant, quand je me regarde je me console, quand je me compare je me désole ! La parole est à M. Jean-François Longeot, pour le groupe Union Centriste.

son dernier rapport, la Défenseure des droits pointe d'ailleurs la mise à mal des droits et libertés de leurs résidents, l'urgence de la crise sanitaire ayant conduit à mettre les Ehpad sous cloche. C'est pourquoi la mise en oeuvre prioritaire de la vaccination au bénéfice des personnes âgées en Ehpad dès le mois de janvier dernier avait suscité légitimement beaucoup d'espoir. Le Président de la République dans son allocution du 31 mars dernier se félicitait d'ailleurs

Les contraintes appliquées aux résidents restent pratiquement les mêmes : confinement et isolement obligatoire en chambre pour une semaine après toute sortie à l'extérieur, maintien d'une seule visite par famille et par semaine, avec une durée limitée à trente minutes. Pourquoi cet excès de précaution ? La situation, vous en conviendrez, devient kafkaïenne. On punit les personnes vaccinées, qui risquent alors de mourir dans la solitude. Le choix de telles restrictions attentatoires à la liberté d'aller et de venir ne peut être laissé à la seule appréciation des directions d'Ehpad, selon la Défenseure des droits.

Cela a nécessité d'apporter dans un premier temps des réponses fortes, sous l'autorité des directeurs d'établissements, dont je salue l'esprit de responsabilité, car personne n'est jamais prêt à faire face à une crise comme celle-ci, qui nous a plongés dans l'inconnu.

La campagne de vaccination en Ehpad est un succès, l'immense majorité des résidents étant aujourd'hui protégée. C'est pourquoi j'ai souhaité, dès le 12 mars dernier, en lien avec le secteur, un protocole allégé, qui est progressivement mis en oeuvre dans les établissements. Très concrètement, un résident bénéficiant d'une couverture vaccinale complète, c'est-à-dire qui a eu ses deux doses, soit l'immense majorité des résidents, ne doit pas être isolé lorsqu'il rentre d'une sortie en famille.

nos forces de l'ordre, incrédules, tiennent le front. Face aux Black Blocs qui s'infiltrent dans les cortèges des manifestations pour piétiner la démocratie sociale, face aux voyous arrêtés qui ricanent, sachant qu'ils seront relâchés le jour même, nos forces de l'ordre, incrédules, tiennent le front. Quand les obligations de quitter le territoire français ne sont pas exécutées, quand vous expliquez que l'immigration n'a rien à voir avec la politique de sécurité, nos forces de l'ordre, incrédules, tiennent le front. Quand elles aspirent à plus de reconnaissance, vous créez une plateforme de signalement des discriminations, qui stigmatise le travail de nos policiers, mais nos forces de l'ordre, incrédules, tiennent le front. Les forces de l'ordre expriment aujourd'hui leur fatigue devant le renoncement de l'État. Une Nation qui ne soutient pas ceux qui se battent pour elle court vers l'abîme. N'importe quoi ! Ma question est donc simple : que comptez-vous faire pour restaurer l'autorité de l'État et réhabiliter ainsi nos forces de l'ordre ?

au commissariat de Rambouillet, depuis vingt-huit ans. C'était l'un des visages de notre police, l'un des visages de ceux qui, au quotidien, protègent. Vous avez raison de le rappeler, il est de notre devoir de protéger ceux qui protègent.

Je compte sur vous pour dire à M. le ministre de l'intérieur que je n'ai fait que relayer la vive inquiétude formulée par les policiers sur le terrain. Comprendre le malaise de cette profession, c'est oser se regarder dans le miroir, un miroir qui renvoie l'image d'un État dépassé, submergé. Nos policiers demandent à leurs enfants de cacher leur profession

La parole est à Mme Martine Filleul, pour le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. la crise sanitaire a mis en exergue les failles de notre système de santé, en particulier le manque de personnel médical, tant à l'hôpital qu'en ville. Les femmes en souffrent plus que les hommes. Ainsi, 30 % des Françaises ne bénéficient pas d'un suivi gynécologique. C'est notamment dû à la quasi-disparition de la gynécologie médicale libérale.

Vous avez d'ailleurs considéré ces professionnels au même titre que les secrétaires médicales, sans même consulter les syndicats concernés. Quel manque de considération à leur égard ! Pourtant, ! Pourtant, ces soignants peuvent contribuer à résorber les difficultés sanitaires, qu'il s'agisse de la lutte contre les déserts médicaux, de la médecine préventive ou encore de l'accompagnement des familles pendant les mille jours suivant la naissance,

C'est ainsi qu'un relèvement du a été décidé, qui montre ses premiers effets sur le nombre des personnes formées et des diplômés. Très concrètement, les effectifs ont augmenté de 23 % entre 2010 et 2020, passant de 18 835

l'organisation des stages universitaires, afin d'orienter davantage les étudiants vers ces territoires. Ce n'est qu'en agissant dès la formation, dès le départ, que nous parviendrons à apporter les réponses pérennes que nos concitoyens attendent.

Voilà plusieurs semaines, la France et l'Europe entière s'indignaient d'une faute protocolaire commise par le gouvernement turc au détriment de la présidente de la Commission européenne.

Monsieur le ministre, ma question est la suivante : que compte faire le Gouvernement pour exiger la libération des prisonniers de guerre arméniens ? Que compte-t-il faire pour que la France reste au rang des grandes puissances et qu'il ne soit pas dit qu'elle a désormais coutume d'abandonner ses alliés

Vous le savez, puisqu'un certain nombre d'entre vous était à Erevan, à l'occasion des cérémonies de commémoration du génocide arménien, avec Jean-Baptiste Lemoyne. Ce dernier s'est rendu auprès des familles de détenus ou de victimes de ce conflit,

Cela aussi, il faut le dénoncer. Pour ma part, je déposerai au Sénat une proposition de résolution invitant à prendre position en faveur de la libération des prisonniers arméniens. Ce serait un signal fort pour nos amis arméniens, mais, c'est clair, ce ne sera pas suffisant. La France ne peut pas rester neutre à ce sujet, car, soyons-en certains, notre inaction et notre faiblesse d'aujourd'hui forgeront notre impuissance de demain. La parole est à Mme Béatrice Gosselin, pour le groupe Les Républicains. Ma question s'adresse à M. le ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Le Royaume-Uni a choisi de quitter l'Union européenne, et le Brexit a été signé le 30 décembre 2020. La proximité du département dont je suis élue, la Manche, avec les îles anglo-normandes est une réalité géographique. Les zones de pêche sont très proches et, depuis janvier dernier, les relations maritimes et commerciales sont mises à rude épreuve. les pêcheurs ont appris à la fin de décembre dernier que les accords de la baie de Granville, qui réglementaient les modalités de pêche, étaient devenus caducs. Les licences d'exploitation affectées aux professionnels de la mer seront désormais délivrées de façon unilatérale par les autorités jersiaises. Vendredi dernier, ces licences sont arrivées pour les bateaux français de plus de douze mètres, et le soulagement a fait place à la consternation, car les laissez-passer n'autorisaient que quelques jours de pêche et imposaient parfois d'autres restrictions. Nombre de petites embarcations, qui ont envoyé les preuves de leur antériorité dans les eaux britanniques, n'ont, à ce jour, pas encore obtenu la licence définitive. Prenons un exemple : un professionnel qui a obtenu, l'an dernier, un permis d'exploitation des autorités maritimes françaises a investi 850 000 euros dans un nouvel équipement ne sait pas s'il pourra pêcher dans les eaux britanniques, la plus grande zone de pêche. Aux inquiétudes des professionnels français, vos services ont répondu, le 3 mai dernier, que l'île de Jersey était souveraine dans sa décision, qui risque d'être irréversible, et que nos pêcheurs recevraient des mesures compensatoires. Mais cette profession, qui représente 2 000 personnes sur la côte ouest, aspire seulement à vivre de son travail ! De Boulogne à Saint-Brieuc, nos pêcheurs subissent des décisions imposées par les Britanniques. Monsieur le ministre, qu'envisagez-vous pour que les professionnels de la pêche ne soient pas les victimes collatérales d'un Brexit qui devait être un accord et qui se révèle être un ultimatum ?

C'est la raison pour laquelle Annick Girardin a pris attache avec la Commission, qui partage d'ailleurs l'analyse de la France sur ces licences, et a demandé que les négociations sur l'accord de la baie de Granville puissent être entamées très rapidement.

J'espère, monsieur le ministre, que vos annonces deviendront réalité, parce que les pêcheurs n'en peuvent plus !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

Depuis décembre 2019, le coronavirus a frappé 150 millions de personnes et fait 30 millions de morts, dont un tiers d'Européens. Même si c'est l'Asie qu'il submerge aujourd'hui, il circule encore très activement en Europe, et nous déplorons encore chaque jour trop de victimes. Le premier outil de prophylaxie étant de limiter les contacts sociaux, la réponse publique à la pandémie a principalement pris la forme de restrictions de liberté, qui ont eu des conséquences de tous ordres, sur l'État de droit et sur notre mode de vie, mais aussi sur l'économie et la croissance et sur la situation sanitaire et sociale. Inédite dans la brève histoire de l'Union européenne, cette pandémie la bouleverse. En remettant en cause la liberté de circulation, elle porte atteinte au coeur même du projet européen. Au vu de la progression de l'épidémie, la présidence croate du Conseil a, du mois de janvier 2020, activé le dispositif intégré de l'Union européenne pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise. Le 6 mars 2020, les États membres de l'Union s'engageaient à apporter une réponse coordonnée à cette crise d'envergure mondiale. La commission des affaires européennes du Sénat en a assuré un suivi attentif. Elle a souhaité que le Sénat puisse en débattre aujourd'hui, au-delà des polémiques vaccinales. Cette crise, comme toutes les autres, mais peut-être plus que les par son impact tous azimuts, agit comme un révélateur ou comme un accélérateur des transformations de l'Union européenne. Par la réponse qu'elle y apporte, l'Union démontre son potentiel, mais aussi ses limites. sa dépendance, qui souligne, en creux, l'enjeu de l'autonomie. La pénurie de masques et de matériel médical en a apporté une preuve flagrante. L'incapacité européenne à produire seule des vaccins l'a ensuite vulnérabilité de l'Union, la pandémie a ouvert les yeux sur les impératifs de résilience et d'autonomie stratégique. Leur portée reste débattue, certains s'inquiétant d'un protectionnisme déguisé ou d'un découplement d'avec l'OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord), mais ces impératifs figurent désormais dans les conclusions du Conseil européen et dans les propositions de la Commission européenne. Ce ne sont pas que des mots : des actions sont aussi menées à la faveur de cette prise de conscience. En décembre dernier, la Commission a ainsi proposé plusieurs textes pour renforcer la régulation des marchés et services numériques et retrouver une souveraineté dans ce domaine. Une ambition industrielle plus large se dessine, afin de doter l'Union de ses propres normes et capacités de production, non seulement en santé, mais aussi dans quatorze écosystèmes industriels ciblés. Même si sa publication a été deux fois reportée, trahissant des tiraillements internes, une mise à jour de la stratégie industrielle européenne est imminente : il s'agit de remédier aux dépendances stratégiques à l'égard de pays tiers, soit en relocalisant certaines productions, soit, à défaut, en sécurisant et diversifiant nos approvisionnements. Un mécanisme permettant à l'Europe de faire face aux pénuries de produits jugés critiques est annoncé, et le rôle des projets importants d'intérêt européen commun sera réaffirmé, y compris au bénéfice du spatial. De même, en matière de politique commerciale, la récente communication de la Commission européenne, publiée au début du mois de mars dernier, atteste d'un changement d'approche : elle insiste sur l'objectif d'une « autonomie stratégique ouverte », qui doit permettre à l'Union de gagner en puissance dans la défense de ses intérêts commerciaux,

Ils ont commandé, surtout au début, des réactions désordonnées dans chaque État membre, par exemple des fermetures de frontières unilatérales. L'année écoulée a toutefois apporté plusieurs preuves fortes de la solidarité qui fonde l'Union. Je pense à l'entraide des soignants ou aux transferts de malades entre pays frontaliers. Je pense à la commande groupée de vaccins par la Commission européenne, qui a permis de garantir à tous les États membres un approvisionnement égal en vaccins, à proportion de leur population.

Je pense surtout à l'éclatante manifestation de solidarité qu'a constitué l'accord politique obtenu en juillet dernier sur un plan de relance européen d'envergure, assis sur un emprunt commun. C'est un pas gigantesque, qui paraissait inimaginable trois mois plus tôt. Apporter un soutien européen à la relance dans tous les États membres est notre intérêt bien compris, mais cela témoigne aussi de la solidarité européenne dans l'épreuve. Le troisième enseignement que nous pouvons tirer ensemble de la réponse européenne à la crise sanitaire est la force de frappe de l'Union, malheureusement atténuée par des pesanteurs internes. De fait, l'Union s'est montrée capable de réagir à la crise : sans compétences en matière de santé, elle a négocié et conclu, presque aussi vite que les États-Unis, plusieurs contrats pour obtenir près de 2 milliards de vaccins. Elle a accéléré ses processus d'évaluation des vaccins et prévoit de se doter d'une agence de recherche biomédicale. Elle propose maintenant un certificat vert pour restaurer la libre circulation dans l'Union. Certes, elle a visiblement sous-estimé le défi que la production de masse d'un vaccin représentait, notamment pour AstraZeneca.

Elle a assuré la circulation des marchandises. Elle a facilité l'accès aux fonds structurels européens. Elle a suspendu- c'est important -le pacte de stabilité et de croissance pour desserrer l'étau budgétaire. Elle a adapté son futur cadre financier pluriannuel pour y intégrer un plan de relance de 750 millions d'euros. L'Union n'a donc pas démérité dans la réponse qu'elle a apportée à la pandémie. Pourtant, elle nous a aussi déçus. J'y reviendrai en conclusion de nos débats, car ces déceptions nourrissent des interrogations de fond sur le projet européen. La parole

vous l'avez rappelé, la pandémie de covid-19 a déclenché une crise inédite pour l'Europe et pour le monde. Cette crise, nous devons encore l'affronter. Il est probablement temps de tirer les premières leçons

à affronter une crise sanitaire, surtout de cette ampleur. Depuis le début de la crise, du chemin a été parcouru. Je veux revenir sur quelques aspects de cette crise multiforme,

: « L'Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises. » Je crois que cette leçon doit encore nous éclairer, au moment où nous essayons de tirer les premiers enseignements

Je veux rappeler que c'est la France et le Président de la République en particulier qui ont pris l'initiative, le 10 mars 2020, d'une première réunion en visioconférence des chefs d'État et de gouvernement pour coordonner au maximum les différents aspects sanitaires et économiques des réponses à la crise dès les premiers jours. Les sommets européens virtuels se sont ensuite multipliés, à une fréquence hebdomadaire, ainsi qu'un certain nombre de réunions des ministres de la santé, tout particulièrement pour essayer de partager l'information et un certain nombre de pratiques, mais aussi d'améliorer autant que nous pouvions le faire la coordination des réponses à la crise. Je veux revenir sur les deux principaux volets qui ont appelé des réponses locales, nationales et européennes à cette pandémie. Je commencerai par les aspects économiques, budgétaires et financiers, parce qu'ils sont éclairants. C'est dans ces domaines que l'Europe avait sans doute, au début de la crise, le plus de compétences et d'outils juridiques et financiers pour agir, et je crois pouvoir dire que, sur ce plan, elle a été au rendez-vous. Elle ne l'avait pas été- en tout cas pas suffisamment ou trop tardivement -lors de la précédente crise financière, qui avait frappé notre continent, voilà une décennie. Elle a été cette fois plus réactive,

la Banque centrale européenne, pour ce qui concerne les États de la zone euro, dont notre pays, et la Commission européenne, s'agissant des règles applicables à notre marché, ont réagi fortement.

considérant, à juste titre, qu'elles n'étaient pas adaptées à la période de crise exceptionnelle que nous vivions. Cette réponse et ce pragmatisme européen ont permis le « quoi qu'il en coûte » qui s'est développé en France comme chez la plupart de nos partenaires.

une situation hospitalière extrêmement difficile, nous avons procédé à des transferts de patients d'une région à l'autre. Près d'un tiers de ces transferts a été mis en oeuvre oeuvre depuis la France vers d'autres pays européens, qui ont offert des capacités d'accueil et, parfois, quelques lits. Je le dis, cette solidarité européenne a sauvé des vies.

L'impatience de nos concitoyens et, parfois, leur ras-le-bol, si vous me passez l'expression, sont parfaitement compréhensibles. Ce sentiment n'est pas spécifique à la France : il traverse, après ces longs mois difficiles, l'ensemble de notre continent.

notre innovation, y compris probablement au tout début de la phase de développement des vaccins, alors que nos partenaires américains, ou même britanniques, ont parfois eu plus d'ambition à cet égard. soit, n'oublions pas que, s'il n'y avait pas eu ce cadre européen d'achat des vaccins, aucune de ces difficultés n'aurait été résolue de manière plus efficace et plus rapide.

Je rappelle que chaque orateur dispose de deux minutes au maximum pour présenter sa question, avec une réponse du Gouvernement pour une durée équivalente. Dans le cas où l'auteur de la question souhaite répliquer, il dispose de trente secondes supplémentaires, à la condition que le temps initial de deux minutes n'ait pas été dépassé.

la levée provisoire des brevets sur les vaccins contre la covid-19, le silence de la Commission européenne est assourdissant. Au nom du secret des affaires, de la défense de l'innovation et de l'efficacité d'une production industrielle censée répondre aux besoins, les multinationales du médicament défendent la préservation des brevets. Or le constat est accablant. Alors que l'on manque cruellement de vaccins- seulement 10 % des Françaises et des Français et moins

notamment parce que Pzifer autorise Sanofi à produire son vaccin. Cet argument ne tient pas une seconde ! Non seulement il faudra patienter jusqu'en septembre prochain, mais, en plus, sans levée du brevet, donc sans accès à la formule du vaccin, on en reste à du simple flaconnage, bien en deçà du savoir-faire des salariés de Sanofi et des besoins de la population. Ma question est simple

Madame la sénatrice, soyons clairs, nous partageons l'ambition, que nous sommes les premiers à avoir portée au niveau international, de faire du vaccin un bien public mondial. La question, au-delà des polémiques, est de savoir comment nous le faisons.

Nous avons décidé de faire du vaccin un bien public mondial, pour permettre que l'on y ait accès. Voilà du concret ! Comment procédons-nous ? Nous examinons toutes les possibilités, y compris en matière de propriété intellectuelle et de transfert de technologies pour créer des capacités de production locale.

de doses de vaccin. Ce mécanisme, qui s'appelle Covax, dispose de plusieurs canaux. La France alloue des moyens financiers à Covax pour cet achat de doses. Aujourd'hui, 42 millions de doses ont été fournies à travers ce mécanisme dans plus de 100 pays, et c'est l'Union

mais vous ne leur en donnez pas la possibilité, parce que vous ne levez pas les brevets. Il s'agit véritablement d'un frein. Vous n'écoutez que les grands laboratoires, qui font des profits colossaux. Cette attitude est criminelle pour l'ensemble de l'humanité ! Je vous demande de réagir, en utilisant la licence d'office, qui existe depuis 1968 et qui n'a jamais été mise en oeuvre.

je salue l'annonce, par la Commission européenne, en février dernier, du lancement de l'incubateur HERA, qui, je l'espère, permettra une lutte plus rapide face à la covid-19. À cet égard, j'attire notamment votre attention sur la volonté de la Commission d'accélérer l'autorisation de mise sur le marché des vaccins.

Cela peut paraître peu, mais nous ne le savons que trop bien, dans la lutte contre la covid-19, chaque jour compte. Comment l'incubateur HERA entend-il remédier à ce problème ? Je m'interroge également sur le mode de gouvernance de la future autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire, elle Il s'agit en effet d'un enjeu majeur, sur lequel il faudra être particulièrement attentif, compte tenu des compétences propres des États membres de l'Union européenne dans le domaine. Une articulation équilibrée entre l'Europe et l'échelon national sera importante,

de recentrer les débats sur l'Europe de la santé et de revoir le partage des compétences entre l'Union européenne et les États membres dans le domaine de la santé., il paraît peu probable que la crise de la covid-19 soit la dernière crise sanitaire d'ampleur mondiale ou paneuropéenne de notre siècle.

Strasbourg comme ville et capitale européennes

les autorités compétentes des États membres de destination, ce qui est logique, les prestataires de services de transport de voyageurs transfrontaliers ...

plateforme numérique qui centraliserait, à l'échelle européenne, les données de santé. Cette perspective soulève les mêmes types de questions- c'est donc un bon exercice.

Le 22 janvier suivant, le Centre alerte sur un risque épidémique élevé. Les conseils de constituer des stocks de tests et de masques FFP2 et FFP3 ne sont pas suivis. Les frontières internes et externes de l'Union européenne sont laissées ouvertes. Il a fallu implorer la Chine pour avoir des stocks. Un an plus tard, le Gouvernement a enfin entendu Marine Le Pen, en fermant les frontières. Vous nous vendez l'Union européenne comme l'échelon efficace pour gérer les défis modernes et internationaux, mais ce sont les États- et en France, les collectivités locales -, qui se sont retroussé les manches pour pallier les carences graves de ce Moloch impuissant : une Union de faiblesses européennes qui aura mis en danger des millions de Français.

contre 34 millions au Royaume-Uni, soit 64 % de sa population, pays qui s'est libéré du carcan européen. C'est une preuve incontestable de l'échec et du naufrage de l'Union européenne, comparé à la puissance d'un État volontaire. La vérité, c'est que nous avons deux mois de retard sur les États-Unis et le Royaume-Uni. Et chaque jour de retard, ce sont des vies perdues. Face à la lenteur du processus de certification des vaccins, l'Allemagne a entrepris de passer commande en son nom propre, tandis que la Hongrie s'est tournée vers la Russie et la Chine avec succès et une avance déterminante sur nous. Josep Borell, haut représentant de l'Union européenne, s'est vu moqué par Moscou et n'a pas réussi à négocier le vaccin russe. L'humiliation est désormais collective. Enfin, l'opacité sur les négociations- contrats, montants et délais -au niveau européen a entaché durablement la transparence démocratique et la confiance des Français dans le vaccin.

La gestion des contrats d'achats anticipés par la Commission européenne doit être évaluée dans ses aspects positifs et négatifs. Ces derniers ont mis en évidence l'importance pour l'Union et ses États membres d'adapter les compétences liées à la santé et de se doter d'outils solides et plus efficaces Je pense notamment à la future Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d'urgence sanitaire. Le travail effectué par la menée par Thierry Breton sur le renforcement de la production de vaccins est loin d'être terminé. Je salue la capacité industrielle européenne déployée, qui devrait permettre une production annuelle de 3 milliards de doses. C'est crucial pour les Européens et pour le reste du monde. La solidarité sera la clé de la sortie de cette pandémie. Nous le savons, car nous y sommes exposés, les variants sont de plus en plus nombreux à circuler. l'Union européenne a présenté l'incubateur HERA, pour se préparer à proposer des réponses rapides face à ces variants et pour anticiper les prochaines évolutions de la pandémie de covid-19. À l'heure où nous amorçons un nouveau déconfinement, nous apprenons que le variant dit « indien » est arrivé sur notre territoire. L'idée qui se dessine est l'évolution du vaccin en fonction des mutations du virus, comme pour celui de la grippe. Monsieur le secrétaire d'État, pouvez-vous nous indiquer comment l'incubateur HERA s'implante dans la stratégie industrielle européenne consacrée aux vaccins à court et moyen terme ?

tout le monde. Voilà plus d'un an, le directeur général de l'OMS nous avertissait que nous étions confrontés à une menace commune, que nous ne pourrions vaincre qu'avec une approche commune. Un an après, nous avons tous appris d'expérience que nul ne peut espérer s'en tirer durablement sans les autres et que l'arrogance de certains dirigeants peut peser plus lourdement sur des libertés et des droits que sur la circulation d'un virus et de ses variants- on pense à l'Inde, au Brésil, à Donald Trump ... Notre pays lui-même n'est pas à l'abri d'une mauvaise trajectoire qui ferait de lui une fabrique de variants La solidarité européenne, c'est le choix d'un mécanisme commun de commande et de distribution des vaccins, ainsi que le choix de l'endettement commun pour engager la relance. On voit les difficultés d'exécution, de cohésion et les tracas- en particulier pour les bassins transfrontaliers. La mise en place du certificat européen, cet été, en harmonisant les règles qui autrement partiraient dans tous les sens, peut contribuer à un équilibre entre santé publique et liberté de mouvement. Le Parlement européen a clairement posé les conditions nécessaires pour cela. Nous sommes particulièrement vigilants sur cette question. La solidarité, c'est aussi et surtout notre capacité à faire toute notre part pour faire respecter les droits de chacune et de chacun dans le monde à être protégé de la pandémie. L'effroyable évolution de la situation en Inde, l'écart vertigineux de vaccination, d'équipements d'urgence de respirateurs entre les pays riches et les pays pauvres montre que l'élan de solidarité mondiale est à la peine. Monsieur le secrétaire d'État, alors que l'Union européenne a bloqué toute demande relative à la levée des droits de propriété intellectuelle sur les vaccins, qui permettrait aux pays émergents de produire eux-mêmes des vaccins génériques, alors que l'accélérateur ACT et le mécanisme Covax assureront au mieux la vaccination de

mes chers collègues, la pandémie à laquelle nous sommes confrontés depuis plus d'un an met l'Europe à rude épreuve, érodant parfois des libertés que l'on imaginait il y a peu de temps encore inébranlables ou intouchables, comme la libre circulation.

Sur ce dernier point, l'accord trouvé en juillet 2020 pour un plan de relance massif est une réussite. Des mesures ont été prises, notamment l'assouplissement par la Commission de l'orthodoxie budgétaire européenne et l'annonce d'un plan d'investissement pour lutter contre les effets économiques de la pandémie. La Banque centrale européenne a, elle aussi, réagi rapidement, en lançant un vaste plan de rachat d'actifs pour alimenter l'économie en liquidités et aider les entreprises européennes mises en difficulté par la pandémie et les mesures de confinement. L'Union européenne et ses États membres ont développé une approche commune et solidaire pour des vaccins sûrs et pour coordonner les stratégies de dépistage dans toute l'Europe. Des coopérations bilatérales transfrontalières se sont également mises en place, comme celle, par exemple, qui a permis le transfert de patients français des hôpitaux du Grand Est vers des pays frontaliers. Afin de mener à bien ces objectifs et d'améliorer les systèmes de santé nationaux, l'Union européenne doit favoriser la coordination des politiques et des systèmes sanitaires entre les États tiers et les États membres, en particulier dans les régions frontalières. Cette pandémie a révélé l'importance de la recherche et de l'innovation dans la lutte contre la crise sanitaire et économique actuelle, ainsi que les possibilités qu'offre ce domaine pour prévenir les vulnérabilités lors de crises futures. Monsieur le secrétaire d'État, quelles sont les actions que mène l'Union européenne en matière de recherche contre le virus et quelles sont ses ambitions pour la suite ? La parole est

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, l'idée du certificat vert numérique a été validée le 29 avril dernier par le Parlement européen à une très large majorité, ouvrant ainsi les discussions avec le Conseil européen. Nous nous en réjouissons. Au regard des difficultés de circulation que la pandémie de covid a pu créer, en particulier dans les régions transfrontalières que je connais bien et dont je suis élue, on peut souhaiter que ce pass facilite les choses, pourvu que les règles soient claires, facilement applicables, non discriminatoires et adaptées aux réalités de terrain. Comme l'ont souligné les débats au Parlement européen, le pass doit apporter une véritable plus-value en matière de circulation. La justification d'une vaccination contre la covid-19, d'un test PCR négatif ou encore d'une immunité à la suite d'une infection me semble offrir la souplesse nécessaire pour assurer rapidement un déploiement relativement large du dispositif, ce que le critère de la seule vaccination ne permettrait pas. Il y a une certaine urgence à mettre en oeuvre ce certificat, non seulement parce que nos concitoyens aspirent à plus de liberté, mais aussi parce que l'économie, notamment le tourisme, en grande souffrance, en a largement le besoin.

confirmez-vous toutes ces orientations ? Si la mise en place du certificat est prévue dès le mois prochain, il faut rapidement dissiper les inquiétudes pour qu'il rencontre l'adhésion de tous. Pouvez-vous nous préciser les précautions qui seront prises afin d'assurer la protection des données personnelles des Français ? La parole

Enfin, votre assemblée aura à connaître du projet de loi qui comporte des dispositions sur le certificat sanitaire mis en place en France, dans ce cadre européen. Vous pourrez donc vous assurer que le processus de vérification et de contrôle des données sera le plus strict possible, comme nous y avons toujours veillé.

d'une Europe qui protège, avec cette idée que l'Union européenne serait un cadre préservé dans une mondialisation qui inquiète. L'Union européenne n'a pas compétence en matière de santé. Toutefois, dans le cadre du marché,

avec une concurrence dommageable entre États membres dont les effets ont compromis jusqu'à l'éthique même des travaux. Toutes ces initiatives sont potentiellement financées au même niveau, avec un maximum de 70 dans certains cas, c'est beaucoup trop ; dans d'autres, cela peut être insuffisant pour marquer un intérêt véritable. Dans ce domaine, la comparaison avec les Britanniques n'est pas flatteuse. À traités inchangés, comment pouvons-nous construire une force de frappe européenne pour conjuguer nos politiques de recherche ?

pour la période allant de 2021 à 2027. Le parent pauvre de notre recherche commune était le soutien à l'innovation en matière de santé. Or, vous avez raison, nous devons accepter de prendre des risques. Financer l'innovation, c'est accepter que des financements publics soutiennent des recherches qui n'aboutiront pas, ou pas tout de suite. Si nous ne l'avions pas fait en matière vaccinale, nous n'aurions pas aujourd'hui des vaccins efficaces le signale, des quatre vaccins aujourd'hui homologués par l'Agence européenne des médicaments- BioNtech, Moderna, AstraZeneca et Johnson & Johnson -, trois sont européens

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, la pandémie de covid-19 a contraint la Commission européenne, comme la plupart des États membres, à changer de paradigme, en acceptant d'abandonner pour un temps les politiques libérales et d'austérité et les règles budgétaires de l'Union plus, après l'accord entre la France et l'Allemagne, elle a préparé et présenté un plan de 750 milliards d'euros, dont une partie est financée par la dette. Cette nouvelle approche face à un défi commun ouvre une nouvelle étape d'approfondissement de l'Union. Cette dette européenne est en fait l'affirmation d'une autonomie stratégique européenne. On ne peut nier les résistances internes face à cette évolution. Dans les États membres, plusieurs parlements tardent à ratifier la décision relative aux ressources de l'Union européenne. À l'échelon européen, la lenteur de la mise en oeuvre du plan européen et son caractère très bureaucratique laissent perplexes nombre d'observateurs. La pandémie contraint de surcroît l'Union européenne à repenser ses priorités et les bases de cette autonomie stratégique. Cela a été souligné pour l'ensemble de l'industrie pharmaceutique et de la santé, mais il ne faut pas oublier des secteurs industriels plus traditionnels, gros employeurs durement affectés par la pandémie, notamment les industries liées au transport.

destine-t-elle si peu de moyens à la rénovation énergétique du logement social ? Enfin, comment justifier, dans le plan France Relance, des mesures structurelles frappant les plus faibles ? Je pense en particulier à la réforme du calcul de l'assurance chômage

d'État, mes chers collègues, la crise du covid a en effet été le révélateur des forces et des faiblesses de l'Union européenne. La force, c'est celle de la solidarité envers les pays défavorisés et, surtout, entre les pays membres, qui ont négocié unis pour éviter une concurrence mortifère concernant l'approvisionnement en équipements de protection personnelle et en vaccins. Toutefois, cette crise a surtout souligné la naïveté des gouvernements, qui ont laissé à l'Europe les clés de la gestion de la pandémie, oubliant que l'Union n'était pas seule au monde et que la concurrence internationale s'exercerait sans pitié pour obtenir les vaccins au plus vite. il s'agit ici non pas de se perdre en conjectures, mais de regarder les chiffres en face. Comment expliquer que les pays de l'Union, avec un poids de négociation de près de 450 millions d'habitants, n'aient pas fait mieux, ou du moins pas aussi bien, que les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore Israël ? Négocier à vingt-sept avec les grands laboratoires aurait dû être une force pour se procurer les produits au meilleur prix et dans les meilleurs délais. Or nous sommes définitivement à la traîne, monsieur le secrétaire d'État, avec un pourcentage de personnes vaccinées deux à trois fois plus faible que dans les pays que je viens de citer. Personne ne peut dire que l'Europe est restée les bras croisés pendant cette période. C'est une réalité, dont nous devons nous réjouir. Mais les gouvernements des pays européens, notamment le gouvernement français, qui devrait pourtant être moteur de l'Union, avec l'Allemagne, n'ont pas su lui donner la souplesse et la réactivité que justifiait pourtant cette pandémie exceptionnelle. Nous devons donc tirer les enseignements de cette situation, pour nous préparer aux futures crises sanitaires qui se produiront immanquablement et nécessairement. Si, pour ce qui concerne la santé, l'Union européenne ne dispose que des compétences réduites que les traités lui donnent et que les États membres veulent bien lui laisser exercer, ne pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d'État, qu'il est crucial de repenser cette politique, en dotant les organes décisionnels européens d'une capacité de réponse audacieuse, rapide et, au besoin, innovante en cas d'événement sanitaire majeur ? La parole est

pourquoi les Britanniques ont-ils gagné un certain nombre de jours et de semaines sur nous ? Pourquoi les Américains ont-ils également pris de l'avance ? Parce qu'ils ont pris plus de risques au départ pour financer l'innovation, les essais cliniques et les dernières phases de développement des vaccins. Il s'agit non pas d'une question de compétences européennes, françaises ou allemandes, mais d'un choix collectif que nous avons fait.

Depuis lors, chaque État membre a fait comme il a voulu, sans coordination excessive avec ses partenaires, même si aucun pays, sauf la France à la fin du mois de janvier, n'a fermé ses frontières à ses propres ressortissants. Depuis maintenant plus d'une année, la liberté de circulation dans l'Union européenne et, singulièrement, dans l'espace Schengen n'existe plus. Chaque pays impose contrôles et conditions d'entrée à ses frontières, parfois même avec des quarantaines pour des déplacements intracommunautaires, même entre voisins. Pour sortir de cette situation, un règlement européen est en cours de négociation. Il créera de fortes discriminations entre ceux qui vivent dans des pays européens où les tests sont gratuits et ceux pour qui les coûts de ces tests dépassent les 120 euros,

Le pass sanitaire a vocation à refaire vivre l'espace Schengen. Mais s'il est discriminatoire et qu'il est systématiquement demandé aux frontières intérieures de l'Union européenne, ne sera-t-il pas une négation de la liberté de circulation ?

monsieur le ministre,

plus souple, qui permet de garantir les contrôles sanitaires. Nous avons toujours été au rendez-vous pour nos ressortissants, y compris quand il a fallu, au tout début de la crise, en rapatrier

de reconnaître comme protecteurs des vaccins qui n'auraient pas été homologués par l'Agence européenne des médicaments. Ce n'est pas une discrimination, mais une nécessité sanitaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous incitons nos partenaires européens à rester dans ce cadre et à n'accepter-

; le rapatriement, c'est pour plus tard. » Je veux bien que le Président de la République écrive à tous les Français de l'étranger pour dire que l'on s'est occupé d'eux, mais ils ont tout de même eu, pendant un an, l'impression d'être largement abandonnés et bloqués à l'étranger. Néanmoins, tel n'était pas le sujet

monsieur le secrétaire d'État, mes chers collègues, les Européens ont confié il y a quelques mois à la Commission européenne le soin de négocier des contrats d'achats anticipés de vaccins. Cette stratégie a permis d'éviter une concurrence néfaste entre États membres pour l'acquisition de vaccins ; elle a aussi révélé les faiblesses de notre continent. Alors que les États-Unis investissaient dès le début de la pandémie dix milliards de dollars dans la recherche et le développement de vaccins, l'Union européenne ne mobilisait qu'un tiers de cette somme. L'Europe a aussi été plus lente, en concluant ses contrats d'achats anticipés en juin 2020, alors que les Américains les avaient déjà signés en février. Par ailleurs, la Commission a fait le choix d'opter en priorité pour des vaccins qui seraient produits sur le territoire de l'Union, comme AstraZeneca ou Sanofi-GSK, au détriment de vaccins plus prometteurs sur le plan scientifique, comme Moderna. À trop vouloir obtenir les prix les plus bas possible, la Commission n'a sans doute pas suffisamment encadré les délais de livraison, en s'assurant que les entreprises seraient en mesure d'honorer les commandes. À ce propos, la Commission européenne a annoncé le 26 avril dernier qu'elle allait saisir la justice à la suite des retards de livraison de la société AstraZeneca. Le groupe pharmaceutique promet déjà de se défendre fermement, estimant avoir respecté le contrat noué avec Bruxelles et faisant valoir qu'il avait d'autres contrats à honorer avec le Royaume-Uni, où le vaccin a été autorisé un mois plus tôt que dans l'Union européenne. Quoi qu'il en soit, cette société

Merci

de justifier d'une vaccination contre le covid-19 ou d'un test PCR négatif, mais également d'une immunité à la suite d'une infection. Si le but affiché est d'obtenir un cadre européen harmonisé permettant de circuler librement au sein de l'Union européenne, certaines ambiguïtés et questions demeurent. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez répondu à

les États membres auront toujours le droit d'ouvrir leurs frontières aux personnes non vaccinées ou de ne pas exiger de test négatif. Le certificat ne devrait pas empêcher les pays d'imposer les restrictions qu'ils souhaitent, en particulier Enfin, si ce passeport est présenté comme n'étant destiné qu'aux voyages, les organismes chargés de la protection des données alertent sur son utilisation pour accéder à certains lieux tels que les musées ou les restaurants.

Je vous remercie

Nous le savons tous, depuis le début de la vaccination dans les États membres, la question d'un passeport sanitaire permettant aux Européens de circuler sur le territoire de l'Union se fait très pressante. La Commission a donc proposé de créer un document unifié, baptisé « certificat vert numérique ». L'élaboration de ce certificat pose néanmoins des questions juridiques en matière de protection des données et de non-discrimination entre citoyens européens. Malgré des problèmes d'approvisionnement, les campagnes de vaccination suscitent l'espoir d'une possible immunité collective dans les mois à venir. question de la création d'un passeport sanitaire européen par la Commission européenne se pose donc. C'est un sujet qui divise au sein des Vingt-Sept. En janvier dernier, la France avançait ainsi plusieurs arguments pour repousser la mise en place d'un passeport sanitaire. sanitaire. Alors qu'une faible part de la population avait reçu au moins une première dose de vaccin, l'heure était encore à la vaccination et non à la réflexion sur ses conséquences en termes de circulation des personnes.

Devoir attester de son état immunitaire est déjà exigé par de nombreux États. Je pense notamment aux certificats de vaccination contre la fièvre jaune. En France, le Gouvernement a lancé le 19 avril un pass sanitaire, système de certification électronique des preuves de dépistage. L'initiative, pour l'instant limitée aux vols vers la Corse ou l'outremer, est adossée à l'application TousAntiCovid. Il me paraît essentiel que la France, au regard de sa situation géographique en Europe, mais aussi de l'importance du tourisme dans notre économie, soit motrice sur ce sujet.

Il s'agissait non pas d'exclure tout certificat ou pass sanitaire, mais d'en définir les bonnes conditions, au bon moment. Nous étions alors et nous sommes encore dans une phase où la priorité absolue est la vaccination et l'accélération de la campagne de vaccination.

Elle met aussi toutes ses forces à réparer ses errements en attendant que les parlements nationaux autorisent la souscription de l'emprunt commun. L'urgence et la gravité de la situation nous ont peut-être fait oublier une question qui n'est pas si anecdotique : à quoi attribuer l'origine du virus ? Aucune preuve n'a été apportée qui vienne confirmer l'hypothèse d'une transmission du virus entre l'homme et l'animal, et le pangolin semble avoir été innocenté ! Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a pour sa part lancé un pavé dans la mare en reconnaissant, il y a quelques semaines, qu'une piste n'avait pas été « suffisamment approfondie » : celle d'un incident de laboratoire. Cette remarque n'est évidemment pas passée inaperçue ; la communauté scientifique mondiale ne cesse de se mobiliser pour en savoir davantage. Une trentaine de scientifiques internationaux demandaient encore vendredi dernier une enquête indépendante afin d'éclaircir les zones d'ombre du rapport produit gouvernements, dont ceux des États-Unis, du Japon et du Canada, ont déploré, eux aussi, dans une déclaration commune, l'impossibilité pour l'équipe mandatée par l'OMS d'accéder « de manière exhaustive aux données et échantillons originaux Si les experts ont pu accéder au marché de Wuhan et au laboratoire, ils n'ont pas eu accès à ses bases de données, qui contiennent pourtant des milliers de séquences de virus collectées sur la faune sauvage ; surtout, ils n'ont jamais pu mener leurs propres investigations. L'objectif est non pas de dire qu'un incident de laboratoire s'est produit, mais de démontrer rigoureusement que cela n'a pas été le cas et de balayer scientifiquement, le cas échéant, une thèse appréciée des complotistes.

que l'OMS se préoccupe d'approfondir les investigations en Chine sur l'origine du virus plutôt qu'elle rappelle à l'Union européenne qu'elle doit accélérer sa campagne de vaccination, ce qui ne lui avait pas totalement échappé ... Il faudra donc poursuivre cet effort de transparence et d'investigation.

Ces déceptions soulèvent des interrogations fondamentales sur l'avenir de l'Union européenne. Jusqu'où est-elle prête à assouplir ses règles, notamment budgétaires, pour éviter un décrochage avec ses concurrents,

Dans quelle mesure l'Union est-elle déterminée à se donner les moyens d'assurer sa souveraineté industrielle, mais aussi alimentaire ? Enfin, peut-on rendre l'Union aussi réactive qu'un État fédéral comme les États-Unis sans aller vers une intégration supplémentaire ?

Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il m'est arrivé d'être critique sur les dispositifs proposés par l'État pour mobiliser les territoires sur la voie d'une réelle transition écologique. J'ai ainsi pu avoir la dent dure sur cette manie qu'ont les ministres et les gouvernements d'inventer en permanence de nouveaux dispositifs. dernières années, nous avons ainsi d'abord connu les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), mis en place par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, lesquels ont aussitôt été occultés par les appels à projets des TEPCV, les territoires à énergie positive pour la croissance verte promus par Ségolène Royal. Quelques mois plus tard arrivaient les CTE, les contrats de transition écologique, chers à Sébastien Lecornu, qui devaient se transformer, avant même d'être généralisés, en CRTE, les nouveaux contrats de relance et de transition écologique, défendus par le trio forment Jean Castex, Jacqueline Gourault et Barbara Pompili. Reconnaissons que cet empilement ne facilite guère l'action territoriale, qui a besoin de cadres clairs, lisibles et stables pour se déployer Ce préambule étant fait, cette insécurité entretenue de l'action territoriale ayant été dénoncée, je me permettrai de brouiller quelque peu mon image de grognon en déclarant- devant témoins, madame la ministre -que parmi les dispositifs que j'ai énumérés, le CRTE, réellement complémentaire du PCAET, est sans nul doute le plus prometteur et le plus cohérent. Madame la ministre, l'objet de notre débat cet après-midi est donc non pas de clouer au pilori le CRTE, mais au contraire de lui permettre de répondre au défi central de la déclinaison territoriale de la transition écologique, sans laquelle nous ne pouvons tenir aucun de nos grands objectifs environnementaux. Il faut en effet rappeler une nouvelle fois que ces enjeux, notamment climatiques, sont tous liés à notre vie quotidienne, à notre manière de nous déplacer, de nous loger et de manger. Or ce sont d'abord les décisions des élus locaux qui permettent de modifier En cherchant à construire un contrat unique avec les territoires, à l'échelle des EPCI, l'État s'engage à plus de clarté sur les financements qu'il leur apporte et propose de les adosser à un réel projet de territoire intégrant explicitement la transition écologique. C'est l'occasion pour les élus de construire, avec les acteurs de leurs territoires, de véritables projets partagés à l'échelle de l'intercommunalité, échelle qui souffre encore bien souvent d'un réel déficit de fonctionnement démocratique. Il n'y a rien à ajouter au courrier que j'ai récemment reçu de Barbara Pompili, qui évoque « un contrat unique ayant vocation à mobiliser les acteurs d'un territoire autour d'un projet de relance écologique à court, moyen et long termes, dans une approche intégrée de l'ensemble des politiques publiques Mais- évidemment, il y a un « mais » ! -une telle ambition nécessite un projet de territoire robuste et partagé. Or l'État, dans sa volonté de relancer rapidement l'économie, a fixé un délai bien trop court pour la conclusion des CRTE. C'est en effet au 30 juin prochain que doivent être signés ces contrats par toutes les intercommunalités de France, c'est-à-dire moins d'un an après l'entrée en fonctions des nouvelles équipes communautaires, qui ont bien souvent appris à se connaître par visioconférence. Il est donc impossible dans un délai aussi court de totalement assimiler les plans précédents et d'actualiser ou de redéfinir avec les acteurs du territoire, eux aussi derrière leurs écrans, un nouveau projet correspondant au programme des nouvelles majorités municipales. Les élus des territoires sont donc très nombreux à nous alerter sur l'impossibilité dans laquelle ils se trouvent de proposer à l'État des projets finançables entrant dans cette belle logique intégratrice que vantent les circulaires du ils définiront en urgence de nouveaux projets correspondant peu ou prou aux attentes de l'État, mais nous savons bien qu'ils recycleront en général des projets plus anciens, des dossiers sans lien avec une quelconque transition, mais déjà ficelés dans les tiroirs. Nous sommes très nombreux à être aujourd'hui interpellés par des élus qui ne comprennent pas cette précipitation ils sont intéressés par la démarche, mais incapables de répondre à son ambition. Pour préparer ce débat, j'ai envoyé un questionnaire aux communes et aux présidents d'EPCI de Loire-Atlantique, mon département. Ils ont été plusieurs dizaines à y répondre. Plus des deux tiers que, en avril, à deux mois de la conclusion des CRTE, ils n'avaient pas encore engagé de réflexion sur le sujet. Un nombre très important de ces maires nous a même écrit n'avoir découvert que grâce à ce questionnaire l'existence d'un comité de pilotage chargé de l'élaboration du CRTE, voire celle du CRTE et des opportunités

par précipitation l'intérêt même du CRTE. Certes, nous savons qu'il sera évolutif, mais si le cadre de départ est mauvais et qu'il apparaît plus comme un passage administratif obligé que comme une ambition nouvelle, le pli sera pris et il sera bien difficile de revenir de revenir dessus. C'est déjà le cas dans certains EPCI, qui s'affranchissent de tout débat avec l'ensemble des maires de leur territoire et discutent directement avec les préfectures. Si j'étais taquin,

l'État, par les signaux qu'il envoie, montre son attachement à la mobilisation des territoires sur l'enjeu climatique. Cela passe par la valorisation des démarches de PCAET aujourd'hui engagées- c'est un succès ! -dans la quasi-totalité des EPCI. Le Sénat garde en mémoire, mémoire, de façon un peu douloureuse, le refus du Gouvernement de le suivre, malgré un vote quasi unanime dans cet hémicycle lors de l'examen des derniers projets de loi de finances, sur l'affectation d'une part de la contribution climat-énergie à la mise en oeuvre des PCAET ; nous en avons souvent discuté ici.

Mais de 2022 ? Reviendra-t-on d'un coup à 570 millions ? Dans ce cas, seuls les plus agiles et, souvent, les plus dotés en ingénierie auront été servis en 2021, ce qui pourrait se révéler assez désastreux en matière de mobilisation pour la suite. Là aussi, ne serait-il plus plus raisonnable de lisser les crédits du plan de relance sur un temps plus long ? Vous le voyez, madame la ministre, les interrogations sont nombreuses ; mes collègues auront l'occasion d'en formuler d'autres encore dans leurs questions. Je le redis, le CRTE peut être un bon dispositif ; alors, n'en gâchons pas les potentialités par une précipitation liée à un plan de relance qui ne lui est pas intrinsèquement lié ! La parole

de vous remercier de m'avoir invité à débattre avec vous cet après-midi des contrats de relance et de transition écologique. Je remercie tout particulièrement Ronan Dantec et le groupe Écologiste - Solidarités et Territoires de cette initiative bienvenue. Vous le savez, les CRTE ont été annoncés dans la circulaire évoquée par Ronan Dantec à l'instant, signée le 20 novembre dernier par le Premier ministre. Ils marquent un changement d'ambition dans la relation entre l'État et les collectivités du bloc local. Les CRTE marquent tout d'abord la volonté de l'État d'approfondir la méthode contractuelle avec les collectivités territoriales.

Le contrat est une manière de mieux articuler les interventions des uns et des autres sur le territoire. De ce point de vue, le CRTE introduit entre l'État et les collectivités une nouvelle forme de coopération, que nous voulons rendre plus étroite et plus efficace. permet aussi de passer aux travaux pratiques en matière de déconcentration et de différenciation, en agissant de façon mieux coordonnée et dans la durée. Le fait de proposer aux collectivités un contrat n'est pas en soi une nouveauté. Jusqu'à présent, tout le monde contractualisait un peu à sa manière, beaucoup nous demandaient de simplifier et de mettre en cohérence ces multiples contrats. Le CRTE est ce qu'on appelle un contrat intégrateur, il regroupe l'ensemble des contrats qui existent sur le territoire.

Il remplace aussi certains contrats qui existaient jusqu'à présent et étaient arrivés à terme. Je pense aux contrats de ruralité et aux pactes État-métropoles. Tous ces contrats et dispositifs sont mis au service de la stratégie définie et portée par les acteurs locaux. En ce sens, le CRTE est bien plus qu'un contrat : c'est un cadre contractuel. On prend en compte les spécificités du territoire à l'échelle de son bassin de vie ; c'est tout l'enjeu du projet de territoire, un projet stratégique global défini par les accords locaux pour six ans et qui est au fondement de la contractualisation.

de la relance, 2021 et 2022, mais bien durant les six années du mandat municipal et intercommunal. Ensuite, le CRTE est un contrat de relance, car nous souhaitons que toutes les collectivités puissent pleinement bénéficier du plan de relance décidé par le Gouvernement. Gouvernement. C'est le cas des régions, avec lesquelles nous avons signé des contrats de plan qui courent jusqu'en 2027 et comprennent un volet « plan de relance » pour leurs deux premières années. C'est aussi le cas de nombre de départements, qui signent actuellement des accords de relance.

EPCI, mais aux projets de territoire. Tous les projets, qu'ils soient portés en maîtrise d'ouvrage par une commune, par un EPCI, ou par d'autres encore, devront trouver leur place dans les CRTE. Je note que cette nouvelle approche a rapidement suscité l'intérêt des collectivités

ont répondu à notre invitation à élaborer avec l'État un contrat de relance et de transition écologique. Précisons au passage que plusieurs intercommunalités se sont parfois

Dantec, que c'est à Nantes, dans un territoire qui vous est particulièrement cher, que le Premier ministre a signé le 22 janvier dernier le premier protocole d'engagement d'un CRTE en France, lequel fixe les premières orientations et met en place la gouvernance de ce nouveau cadre contractuel. Au fond, pour l'État, le CRTE est le moyen de traduire concrètement et efficacement à l'échelle locale les orientations et les moyens définis à l'échelle nationale. Je n'évoquerai qu'un seul exemple : la transition écologique est une priorité transversale des CRTE. Nous avons d'ailleurs organisé la semaine dernière, avec ma collègue Barbara Pompili, le premier comité de pilotage, en présence des associations de collectivités et des grandes fédérations

Vous l'aurez compris, au-delà de la simplification qu'induit le CRTE, nous recherchons surtout une grande efficacité de l'action publique. À terme, nous allons y gagner, pour les élus comme pour les citoyens.

a aussi vocation à permettre d'aborder tous les thèmes qui intéressent à la fois l'État et les collectivités. En d'autres termes, nous souhaitons que le périmètre thématique de tels contrats soit le plus large possible

les CRTE ont vocation à associer tous les acteurs qui participent à la réalisation du projet de territoire. De nombreux départements et régions s'y sont d'ailleurs intéressés et nous disent vouloir soutenir ces J'ai conscience de l'effort d'explication et du temps que cette démarche nécessite ; je sais qu'elle exige une forme d'accompagnement. J'aurai l'occasion d'y revenir ultérieurement au sujet de l'ingénierie.

est aussi respectueuse de la spécificité des territoires, car ces périmètres ont été déterminés en concertation avec les élus et sont différenciés en fonction des coopérations préexistantes.

mais sur les territoires, elle est souvent encore inconnue au bataillon. Les CRTE devraient aider à lui donner la visibilité qui lui manquait. Mais ses moyens ne sont pas augmentés

J'appelle votre attention, madame la ministre, sur l'importance de cet organisme pour les collectivités, en particulier pour la mise en oeuvre des CRTE. l'ANCT sera-t-elle en mesure d'accompagner les collectivités qui en auront besoin et d'identifier les projets d'investissement vertueux permettant de recourir rapidement aux fonds de la relance ? La parole est à Mme la ministre.

d'euros disponibles. En outre, elle anime une plateforme internet dédiée au CRTE, sur laquelle figurent des ressources utiles pour les collectivités et les préfectures. Nous avons ouvert la possibilité pour les collectivités de recruter

des territoires ruraux (DETR) et la DSIL. Ces allocations directes pour les communes ne risquent-elles pas d'être freinées par l'ajout d'un niveau de décision complémentaire ? L'obligation de passer par des contrats territoriaux pour synchroniser une démarche peut être une bonne idée sur le principe, mais risque d'alourdir la procédure. L'ANCT parle de « territorialisation » de la relance. Nous risquons, de nouveau, un affaiblissement de la maille communale, avec un pilotage recentralisé et regroupé à l'échelon des communautés

Signé pour six ans, il doit regrouper l'ensemble des contrats signés entre l'État et les collectivités. Il s'agit, selon vos déclarations, madame la ministre, « de traduire concrètement l'objectif de différenciation qui doit désormais guider l'action territoriale de l'État Nous ne pouvons que souscrire à cette volonté politique de différenciation territoriale. Il importe de reconnaître enfin le rôle des acteurs locaux et la nécessité de personnaliser et d'adapter les projets aux territoires. Il ne faudrait pas toutefois que cette contractualisation, réalisée dans l'urgence, se résume à une compilation des contrats existants, le véritable objectif étant de faciliter l'action des services de l'État.

Les rôles des départements en matière de transition écologique, énergétique et numérique et des régions en matière économique sont essentiels. Comment comptez-vous les associer à cette nouvelle contractualisation ? N'y a-t-il pas un risque que certains EPCI aient plus de mal à atteindre les objectifs fixés, notamment en zone rurale, où les intercommunalités ne disposent pas forcément de compétences, de moyens et de services adaptés ? Madame la ministre, pouvez-vous nous assurer que les besoins en ingénierie seront satisfaits et que cette nouvelle contractualisation ne sera pas mise en oeuvre au détriment des petites intercommunalités ? La parole est à Mme la ministre.

Le CRTE doit aussi permettre de soutenir les collectivités impliquées dans le tourisme rural, lequel requiert non seulement une montée en gamme des hébergements, mais aussi un travail avec les professionnels afin de promouvoir les activités et les produits locaux et de développer l'e-tourisme. Madame la ministre, voilà ce que les élus locaux souhaitent pour réindustrialiser

pensez-vous pouvoir augmenter les dotations évoquées de façon à être à la hauteur des enjeux ? La parole est

Aujourd'hui, la quasi-totalité des intercommunalités ont engagé un PCAET. Pour rappel, c'est la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a confié aux intercommunalités une compétence exclusive en matière d'élaboration et de mise en oeuvre de ces

à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants existants au 1 janvier 2017. Il doit être cohérent, dans ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, avec les engagements internationaux de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

monsieur Benarroche,

illustre la généralisation d'un nouveau mode de collaboration entre l'État et les collectivités territoriales. Avec le renfort des crédits du plan de relance, cette nouvelle génération de contrats territoriaux vise à accompagner les collectivités dans leurs projets, avec une triple ambition : la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale. Cette nouvelle méthode permet aux acteurs locaux- collectivités, habitants et entreprises -de prendre part, aux côtés de l'État, à un véritable projet de territoire. Les CRTE permettent ainsi aux territoires de faire valoir leurs spécificités, tout en s'inscrivant dans une démarche d'ensemble cohérente. Sur mon territoire, de nombreux présidents d'intercommunalité voient dans le CRTE une véritable opportunité de développement. Ce sont ainsi pas moins de quinze contrats qui ont été signés dans le Haut-Rhin. Toutefois, une préoccupation revient régulièrement lors de mes rencontres avec les présidents d'EPCI. Pour mener à bien ces projets dans la durée, l'engagement de l'État est essentiel et doit se traduire par un engagement financier global, qui assure lisibilité et sécurité pour les collectivités signataires. Il semble que cette dimension

La transition écologique est une nécessité partagée ; elle commande d'évoluer vers des modèles de vie durables et raisonnés dans tous les domaines, y compris celui du numérique. L'ANCT a lancé de nouveaux travaux pour aider les collectivités territoriales à bâtir des feuilles de route numériques dans le cadre des CRTE. En effet, la transition numérique des territoires est aussi en cours ; l'État l'a engagée avec la numérisation des services publics à marche forcée. La transition numérique peut aller à rebours de l'objectif de transition écologique : c'est la problématique de l'empreinte environnementale du numérique. Angle mort des politiques publiques, la transition numérique représente pourtant entre 5 % et 10 % de l'empreinte environnementale de notre pays. Cette part ne cesse d'augmenter, du fait notamment d'une consommation croissante de données 4G, et désormais 5G. En effet, plus des trois quarts de cette empreinte sont dus à l'utilisation des terminaux numériques. Au vu de ces intérêts contradictoires, comment concilier, au moyen des CRTE, la nécessaire transition numérique des territoires qui a été engagée avec la maîtrise de l'empreinte environnementale du numérique ? La parole

de souligner que le Gouvernement a fortement accéléré depuis 2017 la transition numérique de notre pays, dans tous les domaines et dans tous les territoires. Dans le domaine des infrastructures fixes et mobiles, l'année 2020 marque un record puisque plus de 5,8 millions de lignes numériques ont été déployées, soit 19 % de plus qu'en 2019.

L'inclusion numérique est aussi un objectif primordial : chacun doit pouvoir bénéficier d'un accompagnement dans l'accès au numérique, afin que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. Les CRTE peuvent être cet outil d'inclusion. La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Comment les citoyens ont-ils été avertis de cet afflux de crédits au moment de voter ? La plupart des élus municipaux n'ont pas été concertés. Je le répète, les délais de signature sont contraignants et risquent de pénaliser les territoires les moins dotés en ingénierie, ce que vous savez,

les étapes d'une planification stratégique et opérationnelle ? Il faut du concret ! Bruno Le Maire a déclaré : « L'exécution sera un point capital. Nous devons dépenser vite et bien pour avoir des effets concrets sur l'activité. » Or la rapidité semble l'avoir emporté sur la qualité des investissements. Le ministre reconnaît lui-même l'impérieuse nécessité de redéployer « des crédits de projets qui n'avancent pas suffisamment vite vers des projets qui avancent plus rapidement ». Oui ! Conclus pour six années, les CRTE se trouvent pris dans une contradiction manifeste entre les objectifs assignés à la relance et la nécessité de concevoir un plan à long terme pour poursuivre les transitions écologiques et industrielles. Madame la ministre, quels sont les critères communs retenus au titre de la relance et de la transition écologique ? ? Comment pouvez-vous nous garantir, au nom de l'équité territoriale, que les grandes métropoles ne vont pas accaparer l'écrasante majorité des financements de cette nouvelle contractualisation ? La

Globalement, comme l'a dit Jean-Paul Prince, nous soutenons fermement les contrats de relance et de transition écologique. Ils seront l'outil qui nous manquait pour décliner territorialement la relance et les politiques nationales d'aménagement du territoire, en harmonie avec les projets de territoire. Cependant, le concept même de CRTE pose un problème de temporalité, problème exposé de manière un peu caricaturale par l'intitulé du présent débat : « ne pas confondre vitesse et précipitation ».

parce qu'il soulève la question bien réelle de l'articulation dans le temps des politiques qui seront regroupées au sein des CRTE, à savoir une politique de très court terme correspondant au plan de relance, d'une part, une politique de long terme correspond aux projets de territoire, Dans les délais très courts qui leur sont impartis, les collectivités et leurs regroupements pourront-ils identifier les projets de relance les plus pertinents ?

et de leurs équipes dans le projet de territoire. Les contrats de relance et de transition écologique permettront de concrétiser des projets locaux et de donner de l'impulsion à nos ambitions énergétiques et écologiques. Toutefois, je tiens à rappeler notre attachement au dialogue direct avec les élus locaux, qui a été longtemps négligé. Dans mon département, je tiens à saluer la décision de la préfecture d'associer les élus locaux à la construction et à la mise en oeuvre des CRTE. Le calendrier du dispositif me préoccupe. Je m'inquiète d'une juxtaposition de la relance rapide, nécessaire face à la crise économique, et de la relance structurelle, vitale aux ambitions écologiques. Le dépôt des dossiers s'est déroulé dans un temps court, peu efficace pour leur constitution.

En rencontrant des élus sur le terrain, je m'aperçois qu'à ce stade le montant des enveloppes disponibles pour les EPCI et les intercommunalités reste inconnu. Aucun élément chiffré sur les projets déposés n'est disponible. Je m'interroge donc sur la tenue du calendrier et sur le risque que ces contrats de relance n'entraînent une logique de compétition entre les territoires. Madame la ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la présentation des budgets, ainsi que sur les indicateurs utilisés pour évaluer les contrats de relance et leur efficacité ? La parole est à Mme la ministre.

du plan de relance et seront pérennes ensuite. J'en viens aux indicateurs d'évaluation des CRTE. L'évaluation des actions constitue un élément clé du pilotage du CRTE pour la collectivité et l'État.

L'un des grands intérêts du CRTE est de permettre aux collectivités de disposer d'une porte d'entrée unique pour solliciter des aides de l'État et d'offrir une meilleure visibilité aux élus.

également sur les besoins d'appui en ingénierie. Avec des délais contraints, les territoires ruraux ayant peu d'ingénierie auront des difficultés à s'organiser pour monter les dossiers, ce qui risque d'accroître les inégalités entre les territoires, cela a déjà été conclurai sur le problème de la répartition des compétences. Plusieurs actions du CRTE sont engagées par l'EPCI, alors que les compétences concernées sont souvent d'ordre communal : actions en direction des commerces, maîtrise du foncier, réhabilitation de l'habitat des centres-villes ou de la voirie Cependant, les maires ne sont pas toujours associés à l'élaboration des futurs CRTE. Madame la ministre, bien que je considère l'aide territorialisée que constituent les CRTE comme essentielle pour l'économie de nos territoires, je souhaite connaître vos réponses à ces quelques interrogations.

Merci Les contrats de relance et de transition écologique pourraient à moyen terme représenter un outil d'articulation de la transition, entre les stratégies territoriales et le financement des actions. Ce cadre organisationnel renouvelé détient un réel potentiel en matière de lisibilité des contrats territoriaux. Néanmoins, des interrogations importantes demeurent concernant le financement, l'articulation, notamment avec les schémas régionaux et l'ensemble des échelons de collectivités, et le soutien en ingénierie. Sur ce dernier point, madame la ministre, il faudrait cesser de supprimer des postes d'emploi public au Cerema et dans les agences concernées afin de préserver les compétences de l'État en matière d'ingénierie. En effet, depuis 2018 et l'exécution du premier budget voté par la majorité actuelle, le ministère de la transition écologique a perdu plus de 4 000 équivalents temps plein

Pour que les CRTE impulsent une véritable relance écologique, il faudrait renforcer l'évaluation de la compatibilité des projets de territoire avec nos objectifs climatiques. Aussi, madame la ministre, quels indicateurs prévoyez-vous en matière de suivi écologique des projets de territoire retenus, par exemple en matière de diminution d'émissions de gaz à effet de serre, d'économie circulaire ou encore d'innovation sociale avec des partenaires issus de la société civile et de l'économie sociale et solidaire ?

pour rationaliser l'offre et le foisonnement des contrats existants qui obscurcissent l'efficacité des mesures d'accompagnement de l'État en direction des territoires. Certes, il faut agir vite,

vous alerter sur le tropisme de verticalité souvent trop largement prégnant. Le dialogue vertueux entre l'État et les collectivités territoriales doit s'inscrire dans une approche ascendante, tenant compte de la réalité de l'existant et non l'inverse. L'innovation publique locale ne doit pas être découragée par un plan national au périmètre préétabli par l'État.

France Urbaine. Permettez-moi d'insister sur le pilotage de cette territorialisation, qui doit fidèlement traduire la déclinaison opérationnelle des orientations portées par France Relance. Les territoires ont besoin de « sur mesure » et les plus fragiles ne doivent pas se voir souffler les financements par ceux qui seraient mieux outillés.

parole est à M. Stéphane Sautarel. Nous voici maintenant dans le Cantal ... Bâtir une politique contractuelle territoriale pour donner de la lisibilité et du sens à l'action territoriale de nos collectivités et garantir l'engagement de l'État dans la durée en leur direction : qui s'en plaindrait ? Disposer d'une approche différenciée ? Oui, bien sûr répondre de manière conforme aux orientations gouvernementales suscite plus d'interrogations. Attention au syndrome des contrats de Cahors qui n'avaient de contrat que le nom ! Disposer d'une vision territoriale des politiques publiques à conduire et des équipements à réaliser ? Oui, bien sûr Écarter ou presque les communes de la négociation, c'est nier qu'elles constituent le socle de nos territoires et de notre République. Créer un guichet unique, faciliter l'accès aux financements ? Oui, encore

des collectivités. La parole est à M. Didier Mandelli. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, il y a quelques semaines, nous débattions ensemble de la politique d'aménagement du territoire de notre pays, en rappelant que la multiplication et l'accumulation des mesures et des programmes ne traduisaient pas pour autant systématiquement une réelle vision politique. Nous débattons aujourd'hui d'une nouvelle mesure, d'un nouveau contrat qui, en réalité, ne contient rien de nouveau. En effet, les contrats territoriaux de relance et de transition écologique ont pour vocation, selon le Gouvernement, de simplifier la mise en place du plan de relance dans les territoires en regroupant les différents programmes lancés par le Gouvernement comme Action coeur de ville, Petites villes de demain ou France Services. Ce n'est donc pas une nouvelle mesure, mais un regroupement de mesures existantes. Lancés dans la précipitation, ces contrats ajoutent encore un peu plus à la confusion des élus, notamment au regard du calendrier extrêmement serré proposé par le Gouvernement. En effet, les élus ont jusqu'au 30 juin 2021 pour s'accorder sur le contenu de ces contrats, alors que les périmètres viennent juste d'être définis par le Gouvernement en mars dernier.

avant la relance, nous avions déjà accordé des dotations supplémentaires, notamment en

Ma première question porte sur l'articulation des CPER avec les contrats existants. J'ai lu en effet dans la circulaire du Premier ministre aux préfets de novembre 2020 lorsqu'un axe stratégique du projet de territoire correspond à un contrat préexistant au CRTE, ce contrat a vocation à être inclus dans le CRTE. » Dois-je en conclure que les financements

et les CRTE. Sur le site de votre ministère, on lit que l'État et les collectivités s'engageront réciproquement dans le cadre d'accords régionaux de relance et, au niveau infrarégional, dans le cadre de CRTE, pourront être la déclinaison du volet territorial du CPER. Les préfets, dans l'instruction qui leur a été transmise en février 2021 sur l'emploi des crédits de la DSIL,

Or j'ai aussi lu que le financement des CPER doit passer par le volet territorial, désormais nommé cohésion des territoires, qui est facultatif. Que va-t-il se passer pour les régions qui n'auraient pas de volet territorial dans leur CPER ?